M. le président du Sénat a pris acte de la fin de plein droit, à compter du 24 juin à minuit, du mandat de sénatrice de la Sarthe de Mme Nadine Grelet-Certenais. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, elle est remplacée par M. Christophe Chaudun, dont le mandat a commencé aujourd'hui à zéro heure. et républicain, l'examen de la proposition de résolution pour une nouvelle ère de la décentralisation, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain

Ce dimanche aura lieu le second tour des élections municipales, aboutissement d'une compétition électorale où s'affrontent idées et visions. Le premier tour a d'ores et déjà démontré que les formations jugées obsolètes en 2017 ne le sont pas tant que cela peuvent en remontrer à des organisations plus jeunes, réduites pour l'heure au rôle de simple figurant territorial. Si ce scrutin se déroule dans des conditions extraordinaires, il est malgré tout l'une de ces respirations qui font se régénérer notre démocratie locale à échéances régulières ; mentionner cette régularité n'est pas innocent en cette saison d'innovation calendaire Toutefois, quelle portée aurait cette élection, à laquelle les Français sont tant attachés, sans l'acte fondateur de 1982, cette onde de choc qui s'est diffusée sur notre organisation institutionnelle ? Elle n'aurait pas le même sens, ni le vote de millions de citoyens la même valeur démocratique. « La décentralisation est la grande affaire d'un gouvernement de gauche et le maître mot d'une expérience de progrès

du siècle ». Pierre Mauroy l'avait défendue pour libérer une « France asphyxiée par le centralisme », promettant aux Français une « nouvelle citoyenneté » faite d'une plus grande participation.

Bref, la loi Defferre, la bien nommée loi « Droits et libertés », fut une véritable bouffée d'oxygène démocratique et l'amorce d'une période de modernisation des territoires où, d'acteur central, l'État devenait accompagnateur. Ainsi, la décentralisation inaugura une nouvelle façon de « faire République

Certes, les collectivités territoriales ne peuvent pas tout faire, ni compenser à elles seules les mutations du capitalisme qui provoquent l'effondrement des territoires industriels, ni inverser les mouvements de populations, ni répondre à toute l'ampleur du défi écologique. Pourtant, la crise liée à l'épidémie de Covid-19 a mis en lumière les blocages et les lourdeurs de l'État central, quand les collectivités territoriales, c'est-à-dire les élus locaux, ont fait la démonstration de leur réactivité, leur adaptabilité et leur inventivité. Reste que, en dépit de nombreuses réussites, des difficultés demeurent : complexification des modes de gouvernance locale, nouveaux rapports aux territoires induits par une société du mouvement perpétuel, contrainte financière, normes, responsabilité des élus locaux, attentes et exigences toujours plus grandes des citoyens. Par ailleurs, sous deux quinquennats marqués par des orientations politiques différentes, les territoires ont connu, de la loi RCT à la loi NOTRe, une véritable fièvre institutionnelle, dans l'attente d'un hypothétique texte 3D. Les réformes ont mis les élus locaux, notamment municipaux, sous tension. Ainsi, au début de 2019, les maires disaient ne pas vouloir de bouleversement institutionnel. Cette attitude s'inscrivait dans un contexte d'incompréhension avec l'exécutif 80 km/h sur les départementales, suppression de la taxe d'habitation, asphyxie des contrats aidés, contrats de Cahors, sans oublier #BalanceTonMaire. Si les élus locaux sont tardivement revenus en grâce pendant la crise des « gilets jaunes », puis des gestes comme l'adoption d'une loi dite Engagement et proximité, il reste que, à la veille des municipales, seuls 31 % des maires disaient avoir confiance dans la parole du Gouvernement pour la mise en oeuvre des futures réformes locales. Par contraste, à travers de multiples initiatives, les élus locaux encourageaient à tirer toutes les conséquences des réformes précédentes et en appelaient à une confiance de l'État dans ses territoires. Dans un environnement difficile, rendu plus volatil par la crise du Covid-19, il est plus que jamais nécessaire de changer notre manière d'appréhender la décentralisation. Il faut rompre avec le prêt-à-penser en la matière,

Cette nouvelle approche, c'est surtout un retour aux sources des lois de 1982. Le principe en était simple : ce qui relève à l'évidence de la proximité et de l'administration du quotidien doit aller vers le local- en d'autres termes, si la perspective organisationnelle est importante, la finalité l'est bien plus. Il faut faire en sorte que les biens et services publics soient distribués plus équitablement sur le territoire, de façon qu'aucun citoyen ne se sente jamais oublié ou mis à la périphérie. Ce nouveau récit territorial a plusieurs implications, à commencer par un recentrage de l'État sur des fonctions énumérées dans la Constitution, les autres compétences relevant du niveau local.

L'État français est la résultante d'une construction historique ; il en porte les stigmates. Notre État raconte une histoire, dessine une mythologie. C'est un État fort, mais, à l'instar d'une pieuvre à la tête trop grosse et aux tentacules territoriaux trop petits, il souffre de la centralisation dont il a hérité et qui s'est encore amplifiée ces dernières années. Cela ne signifie pas que l'État doive s'effacer devant les collectivités territoriales, ni qu'il faille renoncer au modèle unitaire. En doit sortir d'une logique de vassalisation des territoires pour devenir leur partenaire, ce qui permettra de mettre fin aux doublons inutiles entre État déconcentré et

fait, les dispositifs verticaux d'appels à projets lancés par ces agences court-circuitent régulièrement les services déconcentrés et entretiennent des logiques sélectives. cette redéfinition opérée, il convient d'ajuster certaines compétences pour certaines collectivités territoriales : affirmer le rôle social du département, redonner quelques compétences à la région, comme le service de l'emploi et l'apprentissage, et donner une place plus affirmée aux élus locaux dans la gestion des hôpitaux. En outre, il faut rompre avec une vision trop homogène du fonctionnement des EPCI (établissements doivent faire de même, car, pour paraphraser Hobbes, il n'est pas possible que le territoire soit caractérisé par la guerre de tous contre tous. Nous devons installer une logique horizontale, une logique d'interterritorialité. L'interterritorialité est, d'une certaine façon, le pendant de la subsidiarité : elle doit remettre le citoyen au coeur des vécus territoriaux. Si les institutions sont fixes, les populations, elles, sont mobiles, passant d'une institution à une autre. S'il n'y a pas de continuité, par exemple en matière de transports publics, cela pose des difficultés graves à certains Français. il faut élaborer des pactes interterritoriaux, à l'échelle départementale ou interdépartementale. Ils sont la condition de l'affirmation d'une nouvelle justice spatiale pour tous les territoires, des ruralités françaises aux zones urbaines en difficulté. La même perspective est à l'oeuvre s'agissant des territoires transfrontaliers.

La différenciation est, en quelque sorte, l'aboutissement du processus de décentralisation. Naturellement, lorsque nous parlons de différenciation, nous pensons également aux outre-mer.

mesures fortes, il ne sera jamais possible d'atteindre des équilibres au sein des exécutifs locaux ! Il convient également d'accroître les droits des élus d'opposition, d'assurer la séparation des fonctions exécutives et législatives locales

je remercie Éric Kerrouche et nos collègues du groupe socialiste d'avoir déposé cette proposition de résolution, qui s'inscrit dans la perspective du projet de loi de décentralisation, déconcentration et différenciation. il est important que le Sénat, assemblée des territoires, s'empare de ces sujets et soit force de propositions. La crise sanitaire a bouleversé tous nos repères, notamment financiers ; cela ne veut pas dire que le sujet n'est plus d'actualité, bien au contraire. La décentralisation consiste en un transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales : l'économie est gérée par les régions, le social par les départements. Ces derniers sortent clairement renforcés de la gestion de cette crise, notamment dans les territoires ruraux. En effet, les départements

cinquième branche de la sécurité sociale, consacrée à la dépendance, tout en conservant le budget hébergement. De même, il faut favoriser les départements qui embauchent les médecins salariés, afin de répondre au problème des déserts médicaux par l'action de proximité. La décentralisation nous oblige à articuler clarté et souplesse pour répartir les compétences. Ainsi, l'articulation de la compétence « économie » entre le département et la région pourrait être aménagée

Trois maires sur quatre pensent que le transfert de compétences rigide des communes aux intercommunalités a des conséquences négatives ... Si le département est l'échelle pertinente de l'action locale, notamment dans les territoires ruraux isolés, il peut aussi s'avérer pertinent de déconcentrer l'action de l'État et

perdus en trente ans dans certains territoires. L'agriculture aussi doit être soutenue, notamment dans les secteurs d'élevage, et bénéficier de différenciations de la part de l'Europe et de l'État. Il n'y aura pas de ruralité sans agriculteurs

France Services peut être une possibilité. Le tourisme rural également doit être différencié pour être pérennisé. Je pense notamment à la réhabilitation des hôtels et des villages de vacances. La suppression de l'artificialisation des terres de façon uniforme

par décentralisation et réaliser une déconcentration avec un service managé par un sous-préfet développeur, mais surtout différencier, pour adapter l'action de l'État fort aux spécificités de chaque territoire.

force de propositions pour la décentralisation, la déconcentration et la différenciation. Madame le ministre, le Gouvernement doit prévoir, dans le projet de loi 3D, des mesures pragmatiques et efficaces pour maintenir la vie dans les territoires difficiles, notamment ruraux. Monsieur

de résolution de nos collègues socialistes prend place dans un débat récurrent, où les hésitations alternent avec l'audace. La décentralisation est-elle une complainte, un refrain, une exigence ? Elle est en tout cas une conviction, défendue par le Sénat, l'initiative du président Larcher, mais aussi par le groupe Union Centriste, qui, en septembre dernier, a organisé un colloque auquel vous avez participé, madame la ministre,

Les concepts en débat attirent et effraient en même temps. Nous sortons d'un cycle de réformes territoriales inventives pour certaines, comme la recomposition des régions,

qui a desserré l'étau qui emprisonnait le bloc local. À l'issue de ces lois territoriales, les élus ont exprimé irritation et asphyxie. Parallèlement, la crise sociale des « gilets jaunes » a violemment révélé le sentiment d'abandon des territoires. Quant à la crise sanitaire du Covid-19, elle a révélé à ceux qui l'ignoraient la capacité de mobilisation des collectivités territoriales qui leur ont permis d'inventer des solutions ; elle a manifesté aussi l'efficacité d'un partenariat intelligent entre l'État territorial, représenté par les préfets, et les élus locaux. La vérité d'une République construite sur deux piliers- l'État et les collectivités territoriales -s'impose plus que jamais comme une évidence pour la performance de l'action publique au service de nos concitoyens.

législateur, ayant prévu la passation de conventions locales destinées à tenir compte de la spécificité de situations territoriales, avait mis en place une procédure qui, loin de méconnaître le principe d'égalité, constituait un moyen d'en assurer la mise en oeuvre. Traiter différemment des situations différentes n'est donc pas déroger au principe d'égalité : c'est, au contraire, l'appliquer. La définition du mode de scrutin selon la taille des communes fracture-t-elle la République ? La reconnaissance des spécificités des territoires d'outre-mer et la création de la Collectivité européenne d'Alsace fracturent-elles la République ?

par touches ponctuelles, comme si nous ravaudions ou réparions, par un droit des exceptions. Or la République ne peut pas être une addition d'exceptions. Comment réussir ce que nous appelons de nos voeux dans le respect d'une République une et indivisible ? Il faut une volonté affirmée et constante de l'État, dans un esprit de confiance dans les élus locaux. Il faut aussi changer l'esprit de la fabrique de la loi.

Clarifier les missions de l'État central et de l'État territorial est tout aussi nécessaire. Nous devons construire une ossature d'architecture qui replace la commune au coeur du dispositif, par sa compétence générale. Il faut aussi définir, pour chaque niveau d'organisation, un coeur de métier, en permettant une articulation avec d'autres collectivités territoriales par des délégations ou des contractualisations.

Les territoires ne peuvent s'ignorer, ni les métropoles prospérer en cultivant l'indifférence à l'égard de leur territoire. La récente loi d'orientation des mobilités est un exemple de raisonnement pertinent : elle introduit l'échelle des bassins de mobilité, donc des bassins de vie.

d'une audace décentralisatrice, en confiance avec les élus locaux. Dans cet esprit, nous nous sommes pleinement associés à la réflexion initiée par le président du Sénat, à travers la mission de corapporteur de notre collègue Jean-Marie Bockel. Je salue l'initiative de nos collègues socialistes, qui permet d'ouvrir avec vous, madame la ministre, un débat qui ne saurait tarder. Si nous souscrivons à l'esprit général de la proposition de résolution, nous avons quelques différences sur un certain nombre de mesures.

en soit, depuis quelque temps, nous sommes de plus en plus nombreux à appeler le Gouvernement à prendre conscience qu'il est temps d'ouvrir un acte III de la décentralisation. La crise sanitaire n'a fait que confirmer cette absolue nécessité. Où donc était l'État, devenu obèse, dans la gestion des masques ? Totalement absent Ce sont les communes, les régions et les départements qui ont acheté et distribué les moyens de protection nécessaires à l'ensemble de la population. Dans ma commune, nous avons même dû fournir la police nationale pour qu'elle puisse effectuer ses contrôles

demandé ... Oui, l'État s'est perdu ! À vouloir s'occuper de tout, il ne s'occupe plus de rien, notamment pas d'assumer les missions régaliennes, pourtant sa raison d'être : la politique étrangère et la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le bon fonctionnement de la justice- les derniers rebondissements de l'affaire Fillon ne plaident pas en faveur de l'institution judiciaire. Oui l'État s'est perdu, et il est en train d'envoyer le navire France par le fond, alors que notre pays a un potentiel et des ressources peut-être uniques : un territoire et surtout un maillage local extraordinaires, une histoire, une culture, des savoir-faire que le monde entier nous envie et que nous n'arrivons plus à faire prospérer,

1 000 fois oui, il faut passer à un acte III de la décentralisation pendant qu'il est encore temps, au moment où nous abordons un tournant majeur de notre histoire et où nous devons faire face à la crise économique, sociale et environnementale sans doute la plus grave que nous ayons connue depuis 1929. Ce débat capital sur la décentralisation, chacun en est conscient, ne fait que commencer. Nous n'en sommes pas encore à détailler les mesures et les solutions qui nous permettraient de trouver un équilibre entre la capitale et les régions, entre la métropole et les zones périurbaines, entre la ville et les territoires ruraux, car, avant d'en arriver à ces mesures précises, il faut commencer par se débarrasser de quelques contre-vérités. La première de ces contre-vérités est la confusion entre décentralisation et déconcentration. besoin, dans cette noble assemblée, de rappeler nos cours de droit précisant que la première- la décentralisation - consiste à déléguer des pouvoirs aux assemblées territoriales élues, alors que la seconde- la déconcentration -se contente de renforcer les pouvoirs de l'administration préfectorale dans les territoires, ce dont, bien sûr, nous ne voulons pas. J'ai noté plusieurs fois que le Président de la République, pourtant issu de la plus haute école d'administration, fait souvent la confusion entre les deux, sans doute à dessein, imité en cela par notre ami le ministre délégué aux collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, qui m'a fait sursauter il y a quelques semaines en parlant des maires comme des agents de l'État de leurs fonctions ! Effectivement, les maires sont des agents de l'État en ce qui concerne l'état civil, mais ils sont d'abord les élus dotés de la légitimité du peuple, en première ligne pour pallier les défaillances trop nombreuses d'un État devenu obèse qui n'assume plus ses pouvoirs régaliens. La seconde contre-vérité est liée à l'idée que la taille serait un gage d'efficacité-« » serait « ». C'est peut-être vrai dans l'univers économique, car le regroupement y est source de profit, mais cela n'a jamais été prouvé à l'échelon local. En organisant cet improbable regroupement des régions sur un coin de table, le Président Hollande a cru qu'il arriverait à bâtir des régions à la dimension des allemands. la réalité démontre que les super-régions n'ont généré aucune économie d'échelle et qu'elles peinent à s'imposer à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce que, face à leurs concurrentes allemandes, elles ne disposent ni de la légitimité ni de la palette de compétences décentralisées requises pour lutter à armes égales.

Durain. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, nous sommes très fiers de soumettre au Sénat cette proposition de résolution pour une nouvelle ère de la décentralisation. Cette proposition est en effet le fruit d'un travail de longue haleine que nous avons amorcé il y a maintenant plus d'une année : nous avons auditionné des chercheurs, des associations d'élus ; nous avons revu bon nombre de rapports parlementaires abordant la question nous avons revu des dizaines de promesses passées d'un nouvel acte de la décentralisation ; nous avons relu les travaux sénatoriaux, de gauche comme de droite- il y en a à profusion ! - ; nous avons relu M. Macron, celui du début, qui disait qu'il y avait trop d'élus locaux, qui, plus récemment, a compris l'importance de la démocratie locale ; nous avons organisé des rencontres partout en France, au Creusot, à Villeurbanne, à Lille, à Nantes, et j'en passe.

C'est pourquoi nous avons choisi de parler d'une nouvelle ère. Nous sommes ici, toutes travées confondues, des élus issus de millésimes différents, même s'ils sont tous de qualité. Nous avons suivi certaines étapes

de résolution pose en quelque sorte les fondations de la nouvelle ère de la décentralisation que nous appelons de nos voeux. À une époque où beaucoup prétendent réinventer le fil à couper le beurre, nos propositions se veulent réfléchies, applicables, précises et réalistes. Vous pourrez faire le comparatif avec les propositions des députés LaREM, qui, dans leur partie « territoires », évoquaient lundi une proposition visant à « multiplier des contacts entre les écoles et les entreprises » ou à « accélérer la déconcentration des services de l'État sur le territoire On a connu plus précis ! Je suis d'ailleurs certain que leurs collègues sénateurs les nourriront de réflexions plus abouties. Nous défendons avant tout une vision, non pas clientéliste visant à contenter chaque échelon territorial en distribuant des caramels, Il s'agit de faire en sorte que les compétences de l'État soient clairement définies dans la Constitution, celles des collectivités locales devenant la règle pour tous les autres sujets. Il faut que les collectivités deviennent des acteurs à part entière, non des figurants dépendants des dotations de l'État, qui récupèrent trop souvent de nouvelles compétences sans les moyens financiers nécessaires- mon collègue Didier Marie y reviendra. Nous voulons mettre fin à la multiplication des agences nationales, qui signifie trop souvent le retour à des pilotages à distance centralisés et sectorisés tout en signant un démembrement de l'État territorial. Nous n'avons pas peur de dire que, en matière de développement économique, il faut rendre aux régions le pilotage de la politique de l'apprentissage en leur confiant celle du service public de l'emploi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis le début des années 1980 et le vote des lois Defferre, la décentralisation est l'un des principaux mots d'ordre des politiques publiques- presque une incantation magique ! Les réformes se succèdent depuis que l'organisation décentralisée de la République a été consacrée à l'article 1 de la Constitution. L'activité du Parlement sur ce sujet est permanente et quasiment frénétique, chaque gouvernement souhaitant imposer sa marque et chaque ministre donner son nom à une loi. Après les lois RCT, Maptam et NOTRe, nous attendons le projet de loi 3D, pour décentralisation, différenciation et déconcentration. Nos collègues du groupe socialiste et républicain proposent aujourd'hui de débattre de ce que pourrait être le prochain acte de la décentralisation. À vrai dire, il semble que c'est ce que nous faisons depuis bientôt quarante ans, sans parvenir, en dépit des effets d'annonce et des concertations, à la stabilité de notre organisation territoriale. Cela est même suggéré dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, qui indique que, dans leur grande majorité, les maires ne sont pas « favorables à un nouveau bouleversement institutionnel entre collectivités locales ou en matière de compétences ». indispensable de remédier à cette situation. En tant qu'interlocuteur privilégié des élus locaux, le Sénat doit être un catalyseur attentif. Pensons, par exemple, aux imbroglios en matière de compétence « eau et assainissement L'appel à renforcer le plan de soutien aux collectivités dans le contexte sanitaire et économique actuel apparaît comme une priorité conjoncturelle indéniable, alors que la période de confinement a éprouvé nombre de nos concitoyens. Le « plan de rebond territorial », qui se concentrerait sur la santé ainsi que sur la couverture et l'accessibilité numérique, semble également primordial- c'est même une évidence dans la situation que nous connaissons. Les territoires, en particulier ruraux, souffrent d'inégalités profondes qui les empêchent de profiter des facilités offertes par le numérique. Celles-ci sont pourtant nécessaires pour leur développement économique et leur attractivité. Vous le savez, mon groupe y attache une très grande importance, lui qui est à l'origine de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires précisément pour combattre les ruptures d'égalité dans l'accès aux services publics et aux infrastructures, même si cette ANCT est sortie édulcorée des débats du Parlement. Dans la même logique, l'égalité entre les territoires doit également passer par la lutte contre l'illectronisme- une question chère à Raymond Vall et à mon groupe qui gagnerait à être déclarée grande cause nationale, comme nous le soutenons. Cela étant dit, cette proposition de résolution comprend quelques aspects qui nous semblent plus problématiques. Nous restons très sceptiques- pour ne pas dire opposés -à l'introduction d'une clause constitutionnelle attributive de compétences à l'État. Cela nous semble même antinomique avec la stabilité institutionnelle réclamée par les élus, puisqu'il faudrait une nouvelle fois réorganiser toute l'architecture institutionnelle de nos collectivités. Souvenons-nous également des débats interminables entre 2010 et 2015 sur la clause de compétence générale. Pourquoi vouloir rouvrir ces débats ? L'égalité devant la loi est bien sûr l'une des pierres angulaires de la République. L'organisation décentralisée de la République ne peut et ne doit pas nuire à ses caractères indivisible, démocratique et social, qui reposent largement dessus. Une telle innovation constitutionnelle, conjuguée au renforcement du pouvoir réglementaire local, entraînerait des conséquences qui nous dirigeraient vers un modèle quasi fédéral, dont je ne suis pas certain qu'il corresponde aux aspirations de nos concitoyens. La France est un pays riche de sa diversité et splendide par son unité, une condition décisive de son existence, selon l'historien Fernand Braudel. Par ailleurs, en ces temps de crise où tous- collectivités, agents économiques, acteurs associatifs ou simples citoyens -demandent davantage de l'État, il serait paradoxal d'ouvrir cette brèche. Il conviendrait plutôt de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité de l'État. Les inégalités entre collectivités proviennent aussi de la disparité des tissus économiques, que nourrit le manque d'équipement ou d'infrastructures. Sur ce point, rien ne serait pire que de libéraliser l'autonomie fiscale, au risque de créer une véritable concurrence entre collectivités et de favoriser celles qui sont déjà bien pourvues en valeur ajoutée. Il convient d'abord d'améliorer la solidarité financière et la péréquation indispensable à l'unité de notre nation, unité qui serait fragilisée par la compétence de principe des collectivités territoriales hors matières régaliennes. Cela étant dit, nous sommes aussi surpris qu'heureux de constater que l'échelon départemental, celui de la proximité, retrouve grâce aux yeux des auteurs du texte. Chacun se souvient ici que telle n'était pas leur position lors des débats sur la loi Maptam et la loi NOTRe, car la métropole était vue comme un nouvel eldorado. Pour notre part, nous n'avons jamais varié. Je souhaite enfin évoquer les « pactes interterritoriaux prescriptifs », qui visent à garantir « un accès et une distribution équitable des biens et services publics accessibles en moins de trente minutes aux citoyens du périmètre concerné N'ajoutez-vous pas de la complexité, alors que vous la dénoncez à raison ? La subsidiarité que vous défendez ne suppose-t-elle pas plutôt des espaces de liberté qu'étouffent aujourd'hui le pullulement d'échelons administratifs, leur chevauchement et leurs interactions complexes ? Il ne faudrait pas que cette nouvelle ère de la décentralisation ressemble aux précédentes sous les habits nouveaux de la coopération territoriale. Ces observations constituent autant de réserves que je formule au nom du groupe du RDSE à l'égard de cette proposition de résolution.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, les deux crises majeures que nous venons de traverser- celle des « gilets jaunes », puis la crise sanitaire -ont mis en exergue la demande claire de nos concitoyens d'un retour à la proximité. Si, notamment au Parlement, les propositions faites à l'issue de ces deux crises consécutives peuvent varier, il n'en reste pas moins que le diagnostic, lui, est largement partagé. Il me semble que l'on peut à ce titre dresser deux constats indiscutables. Tout d'abord, les périodes mouvementées que nous avons traversées ont mis en exergue le rôle incontournable qu'ont joué, par leur engagement, nos élus locaux, au premier rang desquels les maires, comme garants du lien social. Ce sont bien eux qui incarnent l'État dans ce qu'on appelle désormais couramment « les territoires Ensuite, elles ont mis en lumière la demande d'une décentralisation plus aboutie. Les Français, notamment les élus locaux, n'appellent pas forcément de leurs voeux plus de décentralisation, mais bien, me semble-t-il, une meilleure décentralisation. Au fond, ce qu'ils nous disent est simple : « Nous voulons plus de services publics, proches de chez nous. » La demande de décentralisation est en ce sens l'aboutissement d'un mouvement de retour à la proximité. Derrière le mot de décentralisation, plusieurs aspects se mélangent : la décentralisation la décentralisation au sens strict, c'est-à-dire donner plus de compétences aux collectivités, mais également la déconcentration, c'est-à-dire les pouvoirs donnés aux services de l'État territorial, ou encore la différenciation, c'est-à-dire, comme vous le dites souvent, madame la ministre, autrement dit la possibilité d'adapter les règles selon les spécificités de chaque territoire. Finalement, on comprend que se cachent bien souvent derrière ce mot presque tarte à la crème de décentralisation des attentes multiples, polymorphes, en 3D. Dès lors, chers collègues, le point de départ de cette proposition de résolution est indéniablement partagé. Tous ici, quelle que soit la travée sur laquelle nous siégeons, nous partageons le diagnostic. Tous ici, nous avons entendu la demande d'un retour à la proximité. Et tous ici, nous partageons la volonté d'affirmer le soutien indéfectible du Sénat à notre République décentralisée. La décentralisation n'est en fait qu'une réalité relativement récente de notre histoire politique et institutionnelle. Loin de moi l'idée de profiter de cette tribune pour donner un cours d'histoire sur la V République et les grandes lois de décentralisation. Il me semblait toutefois nécessaire de rappeler que notre organisation décentralisée, si elle n'est pas parfaite, est le résultat d'une construction récente par vagues. La dernière, pas si lointaine, est la désormais célèbre loi NOTRe. Son souvenir doit être encore frais ... Et douloureux ! ... dans la mémoire de certains de nos collègues socialistes auteurs de cette proposition de résolution qui ont eu l'occasion d'en débattre sur ces travées en 2014, alors que leur majorité soutenait ce texte. Je me réjouis donc, chers collègues, de constater que, comme bon nombre de parlementaires et d'élus, vous admettez que la loi NOTRe demande d'être corrigée. Elle a été adoptée plus aboutie, plus particulièrement, selon nous, au profit des collectivités territoriales de proximité que sont les communes et les départements. Un tel mouvement de décentralisation ne pourrait cependant se faire sans repenser, au moins en partie, l'organisation de l'État territorial. La crise sanitaire a prouvé son organisation reste perfectible- j'ai entendu ces dernières semaines, comme nombre d'entre vous, beaucoup de choses sur le fonctionnement des ARS ... Le couple maire-préfet a plus que jamais démontré qu'il fonctionne. Il nous faudra donc tout faire pour le renforcer. Ce mouvement a d'ailleurs déjà été entamé. La loi Engagement et proximité, examinée dans notre hémicycle il y a quelques mois, a déjà oeuvré en faveur des maires et, plus largement, du bloc communal. L'intuition sur laquelle elle reposait, celle que le bloc communal doit être le premier acteur d'une République décentralisée, est d'autant plus forte aujourd'hui. Mes chers collègues, je l'ai dit, nous partageons amplement le constat qui a fait naître cette proposition de résolution. Notre République décentralisée est perfectible

abordée au détour d'une proposition de résolution. Je crois au contraire qu'une telle question, qui fait résonner les fibres les plus profondes de notre histoire politique, qui touche à l'organisation de ce qui fait notre État- l'État à la française -, mérite un vrai débat et que nous engagions nous engagions toute notre responsabilité en l'examinant et en la tranchant. Ce débat sera sans doute animé, il l'a toujours été- l'éternelle opposition des Jacobins et des Girondins l'a prouvé -, mais il sera essentiel. N'amoindrissons pas notre ambition pour la République en la privant d'un réel débat. Pouvons-nous vraiment affirmer aujourd'hui la position du Sénat sur des questions aussi complexes que l'autonomie fiscale des collectivités, la limitation constitutionnelle des compétences de l'État, la répartition des blocs de compétences par échelon de collectivité, l'évolution des nomenclatures budgétaires, la révision des dotations de l'État, le transfert à la carte des compétences, la création d'un pouvoir réglementaire des collectivités ou encore la participation citoyenne, pour ne citer que ces sujets ? Pouvons-nous vraiment prétendre énoncer notre position sur ces sujets, tous vastes et complexes, dont les implications législatives et budgétaires sont majeures, sans avoir réellement débattu, chiffres à l'appui ? Je ne le crois pas- cela d'ailleurs ne ferait pas honneur à la réputation de sérieux de sérieux législatif du Sénat. Vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche partage la déclaration d'intention de nos collègues qui en appellent à une meilleure décentralisation. Cependant, nous ne saurions accepter de restreindre cette question à une simple proposition de résolution. Notre débat parlementaire mérite mieux. Nous en sommes Nous en sommes persuadés, le Sénat doit être en mesure de jouer pleinement son rôle de chambre de représentation des collectivités territoriales face à cette problématique. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. En Marche est dans l'impasse ! La parole est à M. Jean Louis Masson. Madame

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, si l'on veut réussir la décentralisation, encore faut-il qu'elle soit organisée de manière cohérente. Le cadre institutionnel

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste nous présente une proposition de résolution sur la décentralisation. Il faut reconnaître qu'il y a du travail. Les élus locaux ont traversé une situation inédite en tenant honorablement la barre et au plus près des citoyens. Les crises comme celle que nous traversons révèlent les défaillances de l'État et mettent en avant d'autres acteurs sur le terrain qui n'ont pas pu faire autrement que d'agir avec les moyens du bord. Mais les crises sont aussi des moments d'exacerbation des mécontentements, facilitant les divisions. L'organisation territoriale est le coeur de cible de la réduction de la dépense publique- c'est un peu votre leitmotiv, madame la ministre. Elle est surtout questionnée, parce que le principe constitutionnel de libre administration et d'autonomie fiscale des collectivités est rogné. Les élus ne veulent pas d'un nouveau big-bang territorial. Ils aspirent à plus de stabilité- ce qui ne veut pas dire qu'ils

Je ne vais pas faire l'inventaire des lois promulguées sous le quinquennat de François Hollande et les gouvernements de Manuel Valls, dont les conséquences sont ici pointées. Si nous ne sommes pas d'accord sur de nombreux points, je commencerai par évoquer les aspects sur lesquels nous nous retrouvons.

Nous souhaitons également que les élus locaux ne soient pas traités comme un coût à écrêter et qu'ils bénéficient de davantage de place et de reconnaissance, notamment dans l'édiction des dispositions législatives. Nous nous félicitons du consensus trouvé autour de l'échelon départemental, partenaire des communes et des intercommunalités. Ce consensus marque la fin d'une période durant laquelle son existence était menacée alors qu'il s'agit d'un échelon pertinent de décentralisation, mais

À ce titre, madame la ministre, le décret du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet nous semble être un recul déplorable, révélateur des vices de la différenciation territoriale. Les associations de défense du patrimoine et de l'environnement sont vent debout contre ce décret, qui permet de déroger à des normes protectrices, faisant le bonheur de bon nombre de promoteurs immobiliers. Plusieurs de vos propositions, mes chers collègues, nous paraissent prendre un mauvais cap,

C'est une porte ouverte, nous semble-t-il, au dumping social et environnemental. L'État a un rôle à tenir, même si celui-ci s'apparente trop souvent aujourd'hui à une déresponsabilisation de l'exécutif, et ce sur le dos des acteurs locaux et économiques. Le législateur, pour garantir l'égalité des territoires et des individus, doit fixer des règles claires et applicables partout. Cette vision de la République peut et doit laisser de la place aux élus. Le renvoi au pouvoir réglementaire local peut être envisagé, mais dans un cas précis et seulement s'il ne consiste pas en une régression de la loi. Vous souhaitez, mes chers collègues, consacrer la clause générale de compétence des communes. Nous la défendons aussi, mais nous la défendons à tous les niveaux de collectivités- puisque c'est un principe fondateur de la République -pour permettre à ces d'agir en commun avec l'État, d'autant plus en période de crise. Voilà une vision de la décentralisation démocratiquement forte et solidaire, qui donne les moyens au local de répondre aux besoins de la population, contrairement à la logique de spécialisation à outrance des compétences. Nous avons du mal à suivre nos collègues qui déplorent un repli local, défendent une plus grande coopération, mais, dans le même temps, adulent la différenciation, qui est, à nos yeux- mais c'est le débat -, la mère des inégalités territoriales, de la concurrence et des mouvements identitaires. Notre profond attachement à une République unie, indivisible et protectrice ne peut que nous faire bondir à la lecture de certaines propositions telles que, par exemple, l'inscription de manière limitative des compétences de l'État L'État n'est pas un partenaire : cette vision managériale de la République nous semble dangereuse. Les élus locaux savent bien que, lorsqu'ils récupèrent des compétences,

tous gouvernements confondus, et que la crise rend cette dépense maintenant impossible à assumer. Au lieu de céder à la tentation du moins d'État et, donc, à une plus grande marchandisation des services, demandons plus d'État, une décentralisation synonyme d'égalité des citoyens, indissociable d'une déconcentration proche des élus. État et collectivités sont efficaces ensemble cessons de penser seulement en termes de rationalisation. Les politiques territoriales impliquent proximité, complémentarité des niveaux d'action, avec des intercommunalités au service des communes. Nous approuvons à cet égard vos propositions pour plus de souplesse dans l'organisation des compétences du bloc communal, à partir du moment où cette démarche découle d'un dialogue démocratique. En revanche, nous sommes profondément contre l'avènement d'un État fédéral, composé de grandes régions et de métropoles européennes. Pour résumer, nous n'avons pas eu le sentiment d'examiner une proposition de résolution pour une nouvelle ère de la décentralisation,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 25 avril 2019, en clôture du grand débat national, le Président de la République a annoncé sa volonté d'ouvrir un nouvel acte de la décentralisation. Représentant des collectivités territoriales de la République en application de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est donc tout naturellement aux premières loges pour contribuer utilement à cette nécessaire évolution. Si, là encore, il faut bien se garder de tout jeter par-dessus bord pour tenter d'atteindre les rives d'un pseudo-nouveau monde, force est de constater que de nombreuses erreurs ont été commises. La première d'entre elles est de penser qu'entre l'État-nation et les pouvoirs locaux, c'est surtout une affaire de partage de compétences. Dans le meilleur des cas, cette répartition se fait sur des bases rationnelles : chacun se voit attribuer des compétences en fonction de ce qu'il sait ou peut mieux faire. Il est ainsi plus rationnel de confier l'activité de défense et d'entretien de l'armée à l'État plutôt qu'à un syndicat intercommunal. De même est-il sans doute plus astucieux que la collecte des ordures ménagères soit gérée par un syndicat intercommunal plutôt que par une direction d'administration centrale. Malheureusement, dans beaucoup de situations, le partage des tâches ne s'est pas fait de manière rationnelle, mais selon une succession invraisemblable de hasards, d'opportunités ou de réformes administratives ubuesques. Le résultat est que les Français n'y comprennent plus rien. Aujourd'hui, pour retrouver un tant soit peu de cohérence, nous devons à l'évidence nous appuyer en priorité sur des échelons qui ont démontré leur pertinence et leur solidité face à l'usure du temps et aux diverses crises et réformes bâclées qu'a connues notre société. Nous devons nous appuyer sur ce qui est parfaitement identifié par nos concitoyens. Nous devons capitaliser sur ce qui est le fruit de notre histoire nationale et le fondement même de notre République. Je veux parler bien sûr de la commune et du département. L'un des enseignements forts de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, c'est que le couple maire-préfet demeure, et de très loin, le plus efficace et le plus adapté. Faut-il encore que ce dernier ne soit pas considéré comme un simple agent de fabrique ou un commissionnaire dans le meilleur des cas. Il est absolument nécessaire de renforcer la déconcentration pour rendre l'État plus proche du terrain et mieux adapter les prises de décision aux réalités locales. Au regard de la diversité des territoires, de la singularité de leurs ressources, de leur histoire, la différenciation fait partie des gênes de la décentralisation. Elle doit être affirmée et reconnue, car elle constitue le meilleur moyen de réduire les inégalités territoriales et sociales. Cette vision n'est pas celle d'un État qui serait affaibli ou dépecé d'une partie de ses compétences au profit des collectivités territoriales. Bien au contraire ! Les préfets pourraient devenir, à cette occasion, les référents et les représentants de toutes les agences de l'État.

Mais voilà que le temps passe, et je dois malheureusement conclure mon propos. Je souhaite dire, sans esprit polémique, à nos collègues du groupe socialiste et républicain, qu'un tel sujet aurait, je crois, mérité une approche plus large et moins subreptice. Cela nous aurait sans doute aidés à faire abstraction d'un passé encore douloureux, dont François Hollande, Manuel Valls et Marylise Lebranchu sont l'incarnation même. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains s'abstiendra sur cette proposition

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, si d'aventure certains de nos concitoyens avaient encore besoin d'être convaincus de l'efficacité des élus locaux et des collectivités territoriales pour leur assurer un service de qualité en vue de répondre à leurs besoins, je crois que la crise sanitaire aura achevé de le faire. Le travail des élus de terrain a été unanimement salué : ils ont réagi dans l'urgence, fourni ou fabriqué des masques, organisé le confinement puis le déconfinement, accueilli les enfants à l'école, maintenu un bon fonctionnement des services publics locaux, alors que les directives de l'État se faisaient attendre, quand elles ne les obligeaient pas à composer avec des injonctions contradictoires. L'urgence sanitaire a rappelé que les collectivités savaient faire preuve d'une remarquable agilité pour administrer leurs territoires, malgré les contraintes financières qui leur ont été imposées. À cet égard, notre proposition de résolution appelle le Gouvernement à compenser les pertes de recettes et les dépenses spécifiques des collectivités liées à l'épidémie de Covid-19. Nous demandons, dans le même temps, que le Gouvernement mette en oeuvre, dans les meilleurs délais et avec toute la souplesse nécessaire, le plan de soutien permettant à ces mêmes collectivités de relancer leurs investissements et de contribuer ainsi au soutien du tissu économique local. Plus globalement, nous souhaitons remettre à plat la relation financière entre l'État et les collectivités. Nous demandons en premier lieu l'abandon des contrats de Cahors, carcans budgétaires léonins qui, aujourd'hui plus que jamais, sont en contradiction avec les besoins de solidarité et de relance économique. Nous proposons ensuite, comme le demandent les associations d'élus, l'instauration d'une loi de financement des collectivités territoriales, en cohérence avec le projet de loi de finances, qui fixerait les dispositions financières, budgétaires et fiscales les affectant. Cette loi permettra de mettre fin aux incertitudes des collectivités, de leur donner de la visibilité sur les moyens mis à leur disposition. Cette loi de financement pour les collectivités serait un gage de clarification et de transparence permettant d'identifier toutes les composantes des ressources disséminées

les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement, et de mettre en lumière le niveau de dépenses contraintes des collectivités. La dépendance financière des collectivités aux décisions de l'État s'est considérablement accrue ces dernières années. La suppression de la taxe d'habitation ainsi que son mode de compensation non seulement accentueront la dégradation de leur autonomie, impacteront aussi la dynamique de leurs ressources et auront des conséquences incontrôlées sur leurs multiples dotations. Dans ce contexte, la perspective d'une remise en cause des impôts de production ne peut être acceptable. Nous demandons donc la suspension de cette réforme fiscale pour redonner aux collectivités les marges de manoeuvre dont elles ont impérativement besoin dans cette période ; nous proposons de redéfinir le ratio d'autonomie financière en éliminant de celui-ci les fractions du produit d'impôt national transférées et d'instaurer un ratio d'autonomie fiscale. ailleurs, l'État doit assumer une compensation intégrale et évolutive des transferts de charge. De même, l'impact financier des dispositions normatives qui s'imposent aux collectivités locales doit être mesuré et compensé. Aujourd'hui, les ressources et les charges des collectivités sont totalement décorrélées et les principes mêmes de la péréquation obsolètes. Nous proposons d'engager enfin la révision des valeurs locatives, qui fossilisent les inégalités territoriales, et de réviser l'ensemble des dotations de l'État, au premier rang desquelles la DGF, de manière à garantir à garantir un niveau de ressources minimum, notamment en stoppant la minoration des variables d'ajustement et en renforçant leur rôle péréquateur en tenant compte des inégalités structurelles entre les territoires. De ce point de vue, nous pensons qu'il serait judicieux de déterritorialiser la fiscalité économique en organisant un prélèvement et une redistribution à l'échelon d'au moins une zone d'emploi dans le but de neutraliser les concurrences entre territoires et de favoriser la coopération en ce qui concerne l'accessibilité des usagers aux services et aux équipements. Pour éviter les concurrences parfois exacerbées entre territoires, nous suggérons l'encadrement strict des appels à projets, si ce n'est à court terme leur disparition Enfin, nous souhaitons que le futur cadre financier proposé aux collectivités prenne en compte l'absolue nécessité de la transition écologique et de la soutenabilité environnementale des politiques publiques. L'État ne pourra se passer des collectivités et de leurs connaissances du territoire pour agir face à l'urgence climatique. Les collectivités ne veulent plus être les réceptacles des politiques nationales établies sans concertation avec les élus locaux. C'est au niveau des territoires que se jouent les questions de mobilité, de maîtrise de l'énergie et de rénovation énergétique. Il faut que l'État fasse confiance aux acteurs de terrain et les accompagne. Nous demandons à cet effet la création d'une dotation verte territoriale pour donner aux collectivités les moyens du changement que, bien souvent, elles ont déjà engagé, mais qu'elles ne peuvent poursuivre plus avant faute des marges de manoeuvre nécessaires. Cette dotation pourrait être créée grâce à une réorientation des dotations existantes et à l'addition d'une fraction d'un impôt national existant. Elle serait susceptible d'être abondée partiellement par des placements citoyens de type « livret d'épargne pour la transition locale De manière globale, tous les défis d'avenir de notre pays, qu'il s'agisse de la transition énergétique et écologique, de la recherche d'un nouveau modèle agricole, de la réindustrialisation du pays, de l'approfondissement de la démocratie et d'une plus grande association des citoyens à la délibération collective, supposent un puissant mouvement de décentralisation. C'est la raison qui nous conduit à proposer un changement de paradigme, qui verrait les compétences de l'État limitativement énoncées dans la Constitution, celles des collectivités locales devenant la règle pour tous les autres sujets. Pour conclure, je reprendrai volontiers la formule de François Mitterrand, qui est plus que jamais d'actualité : si « la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire, elle a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire ».

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce débat nous donne l'occasion de nous interroger : de quoi la décentralisation est-elle le nom ?

sur une langue commune instaurée par François I à travers la promulgation de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Bravo ! Tout en harmonisant leurs organisations la traduction d'une sorte de monarchie administrative, nos territoires ont conservé de fortes identités dans leurs traditions, leurs modes de vie, leurs singularités culturelles et économiques. L'histoire tumultueuse de notre pays est marquée par ce jacobinisme, synonyme d'unité nationale et de stabilité politique, par l'identification de la commune et du département, dès 1789, comme les échelons de base de notre administration. Force est de constater que cet ordre des choses était suffisamment solide pour rester en l'état pendant plus d'un siècle et demi, jusqu'à ce vent de décentralisation du XX siècle. Syndicats mixtes, intercommunalités, régions et pays ont successivement vu le jour, sans oublier les nombreuses agences, créant une superposition de strates administratives relativement complexe, répartissant les compétences de manière assez peu lisible pour les profanes et créant de nouvelles dépenses de structure qui, par effet cumulatif, ne sont pas étrangères à la colossale dette publique de notre pays. Bien sûr, ces évolutions avaient du sens et correspondaient à de nouveaux besoins en matière d'organisation, à la reconnaissance d'une gestion de proximité, mais elles ont été trop souvent chamboulées et ont parfois autorisé l'État à se délester de certaines charges. Les auteurs de cette proposition de résolution ne peuvent ignorer les effets de la désastreuse loi NOTRe, totalement inaboutie, fruit de la lubie de quelques-uns, ou plutôt de l'obsession de la majorité politique du moment, dont la seule ligne consistait à défaire ce qui avait été construit durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Avec la suppression du statut de conseiller territorial, ainsi que la fusion à marche forcée des régions et des intercommunalités dans la proportion incroyable de 40 %, François Hollande a saccagé le travail de décentralisation des années 1970 et 1980. En dépit de ce capharnaüm administratif, les élus locaux aspirent aujourd'hui à la stabilité et revendiquent un principe assez simple : pas de nouveau transfert de compétences sans transfert de financement équivalent. Vaccinés par la décision sur les nouveaux rythmes scolaires et leur corollaire, le temps d'accueil périscolaire dans les écoles primaires, ils sont devenus extrêmement méfiants et regardent avec attention l'avenir du dispositif 2S2C introduit durant la crise sanitaire liée à la Covid-19. La confiance envers l'État s'effrite et la colère monte même franchement lorsque le Gouvernement décide de manière unilatérale de retirer une partie de l'autonomie financière des collectivités locales en supprimant la taxe d'habitation ... Eh oui ! ... ou encore en retirant la gestion de l'apprentissage La clarification des compétences est essentielle, avec un cadre général, mais aussi des différenciations possibles, comme le prévoyait le projet de loi 3D, désormais reporté. À l'État les missions régaliennes, si malmenées ces derniers temps, aux exécutifs locaux l'administration et le développement au plus proche des citoyens. Les derniers mois ont illustré, si besoin était, la souplesse et la réactivité des collectivités pour répondre aux besoins urgents des administrés. La clause générale de compétence des communes doit être garantie et la place stratégique des intercommunalités, des départements et des régions doit être renforcée en s'appuyant sur un pacte financier stable,

Le renforcement de la décentralisation, souhaité par les acteurs locaux, peut et doit être mis en oeuvre. Confier à chaque niveau de responsabilité les compétences qu'il sait le mieux exercer paraît évident, mais cela doit s'accompagner d'une démarche courageuse pour chasser les doublons et mettre fin à des compétences tellement croisées qu'elles en deviennent illisibles. Nous parviendrons alors enfin à réduire ces dépenses publiques, qui font notre triste singularité européenne et nous privent de marges de manoeuvre pour passer des intentions aux actes et mener des politiques nationales et territoriales véritablement ambitieuses. Pour prendre un seul exemple, si l'accent doit être mis sur la rénovation des bâtiments, le patrimoine public largement dégradé constitue une masse extrêmement importante de gains énergétiques. Lancer un plan État-région spécifique pour ce secteur est sans aucun doute pertinent pour relancer notre économie et converger vers les objectifs environnementaux que nous ne cessons, là aussi, d'empiler au fil des textes législatifs.

engagement. Ce texte montre à quel point la décentralisation est devenue la forme naturelle de l'organisation de notre République, principe d'ailleurs gravé dans le marbre de la Constitution.

-, ou d'autres serviteurs de l'État au-delà des frontières partisanes. La décentralisation est aussi par essence un processus. À ce titre, elle suscite régulièrement réflexions et propositions, plus encore aujourd'hui, après une crise sanitaire que vous avez tous mentionnée et qui a mis à l'épreuve notre organisation territoriale. Aussi, vos propositions ne manqueront pas de venir nourrir les réflexions en cours. Alors même que les conséquences de la crise sanitaire demeurent perceptibles- ne l'oublions pas -, j'ai la conviction que nous devons rester à l'écoute des événements. À cet égard, peut-être aussi de modestie, monsieur Durain -lorsque l'on évoque les supposées réussites des uns ou les échecs des autres, car ils ont tous eu la volonté de servir au mieux leurs concitoyens.

donc rester à l'écoute des événements, mais garder également à l'esprit que la décentralisation est un sujet finalement assez complexe. Méfions-nous dès lors des réactions hâtives, ayons le courage d'assumer que, parfois,

Cependant, des voix se sont élevées ici et au sein des associations d'élus pour demander un approfondissement de la décentralisation.

reprise du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Vous le savez, j'ai lancé en janvier dernier une série de consultations régionales pour échanger avec les acteurs locaux de tous horizons sur leurs attentes en matière de décentralisation.

Enfin, j'ajouterai peut-être qu'une longue vie d'élue locale m'a donné le temps de méditer quelque peu sur ces orientations : j'ai acquis la ferme conviction- c'est la raison pour laquelle j'ai préparé le projet de loi 3D -que la prochaine étape de la décentralisation n'était pas forcément ou ne devait pas forcément être la copie conforme de ce que l'on avait connu par le passé,

Aussi, mardi dernier, le Gouvernement a transmis au Conseil d'État un projet de loi organique relatif aux expérimentations territoriales. La différenciation territoriale, dont les premiers jalons seront posés dans ce texte, est bien le nouveau visage de la décentralisation. Elle mettra fin à une conclusion binaire,

Dans un pays construit depuis plus de deux siècles sur l'uniformisation, c'est bien sûr une révolution même si, je le dis pour rassurer ceux qui s'inquiètent de l'expérimentation ou de la différenciation,

le projet de loi organique facilitera l'expérimentation et, donc, la différenciation. Le grand historien Fernand Braudel écrivait, non sans admiration d'ailleurs, que « la France se nomme diversité ». C'est cette diversité que nos politiques publiques doivent désormais mieux prendre en compte pour s'y adapter. Il faut affirmer que des réponses différentes peuvent être apportées en fonction de la singularité des situations.

la Collectivité européenne d'Alsace, qui peut désormais exercer des compétences spécifiques et particulières, notamment sur des sujets qui la concernent au premier chef : je pense, par exemple, à l'expérimentation transfrontalière.

mais pour en tirer le meilleur parti et tirer le meilleur parti des situations. C'est pourquoi le fait d'inscrire dans la Constitution ce qui relève du régalien ou non, ce qui relève seulement des compétences locales ou non, n'est à mon avis ni possible ni souhaitable.

La clarification des compétences est, bien sûr, un point important. La loi NOTRe, tant décriée,

Ainsi, nous renforcerons la concorde républicaine pour mieux protéger notre pays à l'avenir, car, depuis son origine, la décentralisation est une manière de préparer la France

Pour cela, a-t-il souligné, nous devons donner « des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies », sans écarter de pistes. Amen ! Face à la crise écologique, face à la crise sanitaire, il est temps que l'État et les collectivités scellent une nouvelle alliance pour remporter la bataille des transitions,

vous le savez, à la suite des concertations menées dans le cadre du projet de loi 3D, nous avons approfondi la décentralisation dans plusieurs domaines la transition écologique, le logement, les transports. Par ailleurs, nous devons tirer les conséquences de la crise sanitaire dans le domaine de la santé et des solidarités. Enfin, c'est une problématique majeure, il nous faut accélérer la réforme de l'organisation territoriale de l'État. Vous avez tous évoqué

accélération pourrait se traduire par un renforcement du mouvement de déconcentration des moyens, des pouvoirs et des agents de l'État. La restauration de l'unité de la parole de l'État dans les territoires, notamment autour de la figure du préfet de département,

! Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explications de vote.

et républicain, la discussion de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes du Covid-19, présentée par Mme Victoire Jasmin et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à Mme Victoire Jasmin, auteure de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, dans cette France du 25 juin 2020, qui commence progressivement à panser les plaies de cette terrible pandémie, la proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter est un texte attendu et espéré par beaucoup. Mes premières pensées sont évidemment pour les victimes de la Covid-19 et leurs familles. Je tiens également à associer à nos travaux mes collègues du groupe socialiste et républicain,

remercie pour les amendements proposés afin d'améliorer le texte initial. Ce texte, rédigé durant les heures les plus tragiques de la propagation de l'épidémie de la Covid-19 en France et partout dans le monde,

Bien sûr, au fil des jours, les applaudissements à vingt heures et les manifestations de gratitude envers les premiers de corvée

aux agents de la RATP. Je pense aussi aux bénévoles de la réserve sanitaire, et à tant d'autres qui se sont mobilisés pendant le confinement.

Face aux risques accrus de contagion et de morbidité associés au coronavirus SARS-CoV-2, nous avons en urgence dû adopter des mesures exceptionnelles de confinement, afin de mettre à l'abri le plus grand nombre d'entre nous. Ces mesures de salubrité publique nous ont permis d'épargner de nombreuses vies, et, même si le bilan des décès suite à l'infection reste trop lourd, nous pouvons collectivement nous féliciter de la réussite de ce confinement. Pour autant, certains travailleurs et bénévoles ayant poursuivi leurs activités professionnelles ou associatives

Parmi les malades de la Covid-19, peu sont des professionnels qui ont dû maintenir leurs activités pendant le confinement. Heureusement, l'immense majorité de ces professionnels ont été atteints d'une forme bénigne, parfois passée totalement inaperçue et sans aucun impact sur leur état

Comme cela fut annoncé par le ministre des solidarités et de la santé, le 23 avril dernier, certains pourront prétendre à des réparations au titre de la maladie professionnelle. Il est heureux qu'à l'approche de l'examen de cette proposition de loi le Gouvernement se soit enfin décidé à accélérer la publication des ordonnances et décrets permettant cette reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle pour les soignants. Mais cette avancée réglementaire ne permettra pas de reconnaître les services rendus à la Nation par tous ceux qui ont travaillé.

et de la Direction de la sécurité sociale. Ces entretiens ont mis en lumière la nécessité d'instituer un processus d'indemnisation simplifié et équitable de tous les travailleurs ou bénévoles qui, par obligation, auraient été exposés à un risque accru de contamination pendant le confinement. Il va sans dire que le fonds qu'il vous est proposé de créer ne se substitue pas au régime d'indemnisation des maladies professionnelles. Il en est clairement complémentaire ! D'ailleurs, opposer les deux mécanismes

parfois de soldats exposés au risque de contamination, à un moment, faut-il le rappeler, où la France manquait cruellement de masques. Je suis certaine que le Gouvernement a tiré les premières leçons

et des critères objectivables, afin de permettre la réparation intégrale des préjudices subis par un nombre limité de personnes, professionnels ou bénévoles ayant dû poursuivre leurs activités pendant le confinement pour que nous soyons là, aujourd'hui, et qui en

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la création d'un fonds d'indemnisation au titre d'une contamination par un agent pathogène à transmission respiratoire peut surprendre. Ce serait en effet une première. J'entends, bien entendu, les interrogations légitimes de plusieurs de mes collègues sur l'opportunité de créer un précédent, qui risquerait de fragiliser notre système assurantiel de réparation des risques professionnels. Ce système repose sur la responsabilisation des employeurs dans la protection de leurs salariés, protection qui s'est avérée difficile à garantir face à une maladie infectieuse ayant largement circulé dans la population générale, bien au-delà des seules situations professionnelles. Je voudrais néanmoins rappeler l'esprit de cette proposition de loi, déposée par notre collègue Victoire Jasmin, que je salue. Ce texte a pour objectif essentiel de répondre à une situation parfaitement inédite. Il vient reconnaître l'engagement professionnel et bénévole de nombreux de nos concitoyens pendant la phase aiguë de l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité de services indispensables à la vie de la Nation. Dès le début de l'épidémie, les soignants et personnels d'établissements de santé et médico-sociaux se sont mobilisés pour prendre en charge les malades. À cette occasion, ils ont été exposés à un risque accru de contamination par le SARS-CoV-2, d'autant que les équipements de protection individuelle faisaient défaut. C'est la raison pour laquelle le ministre des solidarités et de la santé a annoncé la mise en place, en faveur des soignants, d'un dispositif de reconnaissance automatique comme maladie professionnelle de leur contamination. Toutefois, les contours de ce dispositif n'ont pas été précisés : nous ne savons pas s'il intégrera les personnels administratifs et d'entretien de ces établissements, et il devrait vraisemblablement se limiter à une réparation forfaitaire. Par ailleurs, pendant le confinement, au-delà du soin, d'autres secteurs d'activité ont continué de fonctionner afin de répondre aux besoins essentiels de la Nation. Je pense aux premiers secours, aux ambulanciers, aux forces de sécurité, aux personnels de l'éducation nationale et des crèches qui ont accueilli les enfants de soignants, aux services d'aide à domicile, aux services de propreté et de salubrité publique, aux salariés des pompes funèbres, aux salariés de la grande distribution, des transports, de la logistique et de la livraison, du secteur postal ou encore aux salariés des abattoirs ... La réalité est la suivante : ces nombreux travailleurs et bénévoles, qui ont dû poursuivre leur activité en dehors de leur domicile pendant le confinement, ont été exposés à un risque accru d'infection par le coronavirus. Certaines de ces personnes ont développé des formes graves de la Covid-19, qui ont pu donner lieu, notamment à l'issue d'une hospitalisation dans un service de réanimation, à des séquelles invalidantes ou incapacitantes, telles que des atteintes respiratoires, neurologiques, cardiaques ou dermatologiques, ou ont pu conduire à des décès. Or quels sont les recours s'ouvrant à elles pour obtenir une réparation juste de leurs préjudices, en reconnaissance du service rendu à la Nation ? À tout le mieux, elles devront s'engager dans une procédure longue de demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, avec un risque d'inégalités de traitement et, donc, de contentieux.

proposition de loi vise à instituer un processus d'indemnisation intégrale simplifié et équitable de l'ensemble des personnes qui auraient été exposées à un risque accru de contamination pendant le confinement, au-delà des seuls personnels soignants. Comme c'est déjà le cas pour les victimes de l'amiante, cette réparation intégrale pourrait, le cas échéant, venir compléter la réparation forfaitaire obtenue par les travailleurs par la voie des tableaux de maladies professionnelles nouvellement créés ou des CRRMP. Afin d'acter le lien entre l'indemnisation et le service rendu à la Nation par des personnes qui n'ont pu rester confinées, j'ai présenté en commission plusieurs amendements destinés à circonscrire tant le champ des bénéficiaires du fonds que son horizon temporel. J'ai notamment proposé de définir les éléments qui permettront d'établir une présomption irréfragable de contamination en milieu professionnel ou bénévole, dans le souci d'alléger la charge de la preuve pesant sur les victimes. Ces éléments auraient pu reposer, d'une part, sur une liste d'activités professionnelles ou bénévoles ayant été exposées à un risque accru de contamination et, d'autre part, sur des critères objectivables permettant de présumer, avec une assurance raisonnable, une contamination en milieu professionnel ou bénévole. Ensuite, afin de consacrer le caractère exceptionnel du dispositif, j'ai proposé à la commission de fixer une borne temporelle au risque d'exposition professionnelle ou bénévole à la contamination justifiant une indemnisation intégrale.

Cette période aurait débuté le 16 mars 2020, date de mise en place du confinement, et aurait pris fin à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020. Enfin, s'agissant du financement du fonds, j'ai eu le souci de ne pas le faire reposer uniquement sur une contribution de la branche AT-MP, dont la logique assurantielle est régulièrement mise à mal. L'exposition au virus d'agents de l'État et l'indemnisation des ayants droit de personnes décédées plaident en effet pour une mobilisation de la solidarité nationale par un engagement financier de l'État. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission que le financement du fonds s'appuie également sur une contribution de l'État. La commission des affaires sociales n'a pas adopté ces propositions de modification, qui, à mon sens, auraient garanti la crédibilité et le caractère opérationnel d'un dispositif qui entend répondre à une situation, je le répète, exceptionnelle. La commission a en effet estimé que, en l'état des connaissances scientifiques parcellaires sur les effets à long terme sur la santé du virus, les conditions n'étaient pas réunies pour instituer un fonds d'indemnisation. Pour autant, la majorité de la commission des affaires sociales a clairement affirmé que son abstention sur le texte en commission ne vaudrait pas adhésion en séance publique. Le texte qui vous est donc soumis en séance est essentiellement celui de la proposition de loi initiale, dont les articles n'ont pas été modifiés, seul l'intitulé du texte ayant fait l'objet d'une rectification rédactionnelle. Bien que mes propositions de modification n'aient pas été retenues en commission, je vous invite, à titre personnel, à adopter ce texte. La parole est à M. le secrétaire

Madame la présidente, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la crise sanitaire que nous venons de vivre est, à bien des égards, inédite : inédite par sa fulgurance et sa diffusion- jamais un virus n'avait circulé aussi vite sur l'ensemble de la planète inédite par sa mortalité auprès des plus fragiles d'entre nous, inédite, enfin, par la mobilisation que nous lui avons opposée. L'ensemble de nos forces sanitaires se sont mobilisées, en première ligne face au virus, sans faillir. Le pays a ainsi continué à vivre grâce à ces travailleurs de « deuxième ligne », pour citer le Président de la République : agriculteurs, éboueurs, enseignants, chauffeurs routiers, manutentionnaires, hôtes et hôtesses de caisse, travailleurs sociaux, pas exhaustive -les maires et les élus locaux, que votre chambre, mesdames, messieurs les sénateurs, représente si bien. Vous avez raison, madame la sénatrice Jasmin, les conditions que l'épidémie nous a imposées pour les funérailles des victimes du Covid-19 ont été douloureuses pour les proches et pour les familles. L'ensemble des Françaises et des Français se sont mobilisés face à cette épidémie. La crise sanitaire n'est d'ailleurs pas achevée, et les actualités internationales nous montrent qu'il nous faut rester vigilants partout, y compris sur notre territoire. Pourtant, à la crise sanitaire s'ajoute maintenant le risque d'une crise socio-économique. Nos concitoyens ont fait face, il est donc normal qu'ils demandent de la protection face à cette crise. Dans l'urgence, le Gouvernement y a répondu activité partielle généralisée, primes au personnel soignant, plan de soutien aux secteurs sinistrés, allocation exceptionnelle pour les plus fragiles. Nous sommes aujourd'hui dans une seconde phase, avec le Ségur pour le monde de la santé, mais aussi le soutien aux salariés et aux entreprises et la préparation du plan de relance de l'activité. Cette proposition de loi déposée par Mme la sénatrice Victoire Jasmin et ses collègues du groupe socialiste et républicain vise à indemniser les personnes qui ont été touchées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle prévoit une indemnisation intégrale de toutes les personnes atteintes du Covid-19 ayant été en contact avec des personnes contaminées ou des objets susceptibles de l'être dans le cadre de leur activité professionnelle ou bénévole, ainsi que leurs ayants droit. la sénatrice, partage votre attention sur ce sujet sensible, éminemment complexe. Je connais la difficulté des personnes atteintes du Covid dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi que celle de leurs proches. Selon cette proposition de loi, il reviendrait au demandeur de justifier de sa contamination dans un cadre professionnel. Une commission médicale indépendante constituée au sein du fonds se prononcerait sur le lien entre la contamination et la pathologie. Mesdames, messieurs les sénateurs, la prise en charge des travailleurs atteints du Covid-19 dans le cadre professionnel est indispensable. C'est une préoccupation majeure du Gouvernement. Tout d'abord, nous souhaitons apporter une attention particulière aux soignants- cela a été dit par Mme la rapporteure et par Mme la sénatrice Jasmin.

Nous avons un devoir : faire en sorte que les soignants ayant contracté le Covid-19 après avoir soigné des patients atteints puissent obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle et une indemnisation en cas de séquelles et de décès. S'agissant de ces travailleurs de première ligne, c'est la moindre des choses. Pour les autres travailleurs contaminés dans le cadre de leur activité professionnelle, nous voulons une indemnisation facilitée. C'est un objectif que je partage avec vous. Madame la rapporteure, je ne partage cependant pas l'idée de créer un fonds d'indemnisation dédié, ce qui est le coeur de cette proposition de loi. Nous parlons de risques professionnels, nous parlons de travailleurs notre sécurité sociale dispose d'une branche dédiée à ces questions, la branche accidents du travail et maladies professionnelles, dites AT-MP, que vous avez vous-même évoquée dans votre propos. Cette branche est la plus ancienne de notre système de protection sociale. Elle est gérée par les partenaires sociaux, et c'est d'ailleurs un pilier de notre démocratie sociale. Enfin, cette branche fonctionne bien. Elle est tout à fait apte à cette mission. À l'inverse, je le crois, créer un fonds serait un dispositif lourd et complexe. Il faudrait prévoir une expertise individuelle sur chaque dossier, ce qui serait aussi une source de nombreux contentieux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne crois pas que cela soit l'intérêt des victimes. Ce que le Gouvernement propose, c'est de mettre en place un système de reconnaissance simplifié et rapide. Il se traduira par des décrets qui seront présentés très prochainement aux partenaires sociaux, comme le prévoient les textes en vigueur. Nous allons donc créer un tableau de maladies professionnelles dédié. Il permettra à tous les soignants atteints d'une forme sévère de Covid-19 de bénéficier d'une reconnaissance en maladie professionnelle. Comme cela m'a été demandé, je veux concernera tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux, tous les personnels non soignants travaillant en présentiel dans ces structures, toutes les personnes assurant le transport et l'accompagnement des personnes atteintes du Covid-19. Les professionnels de santé libéraux bénéficieront de cette reconnaissance dans les mêmes conditions que les autres soignants. Pour les travailleurs non soignants- je crois que c'est notre objectif commun -, la procédure sera facilitée. En lieu et place des comités régionaux, un comité national dédié au Covid-19 sera constitué ; il assurera un traitement homogène et rapide des demandes. La reconnaissance des maladies professionnelles est importante, vous le savez. Elle permet une prise en charge des frais de soins à hauteur de 100 % des tarifs d'assurance maladie, une prise en charge plus favorable des indemnités journalières et une indemnité en rente ou en capital en cas d'incapacité permanente. Une rente est versée aux ayants droit en cas de décès, s'élevant à 40 % du salaire de la victime pour l'époux survivant et à 25 % pour chaque enfant à charge, jusqu'à leurs 20 ans. C'est une indemnisation importante pour les victimes, dans un cadre simplifié et efficace, avec une prise en charge adaptée à l'origine professionnelle de la maladie. Avec ces mesures, le Gouvernement entend atteindre l'objectif de votre proposition de loi. Je veux maintenant aussi parler de financement. Le Gouvernement ne souhaite pas faire porter la charge de l'indemnisation sur les employeurs directement concernés. Ce serait un non-sens pour ces entreprises qui se sont mobilisées pendant la crise. Nous souhaitons donc mettre en place un dispositif de mutualisation, puisque la cotisation AT-MP comprend une part mutualisée entre tous les employeurs. C'est bien une question de solidarité nationale et, là aussi, je crois que nous pouvons nous retrouver. Cette part sera prise en charge par l'État pour les professionnels de santé libéraux qui ne bénéficient pas d'une couverture AT-MP. Madame la rapporteure, je souhaiterais enfin souligner les risques de précédent que constituerait la création d'un fonds dédié. J'ai entendu dans votre propos liminaire que vous n'aviez pas souhaité les éluder, ce dont je vous remercie. Une indemnisation en dehors de la logique de la branche AT-MP ouvrirait le sujet sur l'ensemble des maladies professionnelles. Cela mettrait en danger les fondements de la branche, qui permet une reconnaissance rapide et facilitée aux travailleurs en contrepartie d'une indemnisation déterminée. Comment justifier qu'une personne ayant contracté le Covid dans un cadre professionnel soit mieux indemnisée qu'une autre atteinte d'un cancer professionnel ? La différence de traitement ne se justifierait pas, et ce sont donc les principes de la branche AT-MP qui seraient ébranlés. Rappelons que cette branche fait l'objet d'un consensus social de très longue date. Elle permet une indemnisation rapide de plus de 650 000 accidents du travail et de 50 000 maladies professionnelles par an. Madame la rapporteure, vous l'aurez compris, je partage pleinement votre objectif, comme, je le crois, l'ensemble de vos collègues sénateurs et sénatrices. Les Françaises et les Français qui ont permis au pays de tenir méritent notre reconnaissance. Pour celles et ceux qui ont été victimes du Covid-19, nous devons être au rendez-vous. Vous l'aurez compris aussi, le Gouvernement est attaché à la sécurité sociale et à la branche AT-MP, qui permettent d'indemniser les travailleurs touchés dans le cadre de leur activité. C'est pour cela qu'il propose d'agir par décret, rapidement, et dans le respect de la démocratie sociale. Il s'agit d'un choix de cohérence : nous le devons à tous ces travailleurs et à leurs familles. Vous pouvez compter, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, sur mon engagement et celui du Gouvernement pour mettre en place cette indemnisation dans les meilleurs délais.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de Mme Victoire Jasmin portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19. Avant toute chose, mes pensées se dirigent vers celles et ceux qui ont perdu un proche atteint par ce virus, mais aussi vers les familles dont un proche souffre encore aujourd'hui de ce mal. J'adresse mes pensées les plus solidaires aux pays qui font face en ce moment même au pic épidémique ou à une reprise de l'épidémie sur leur territoire. Force est de constater que cette pandémie s'est propagée à une très grande vitesse à travers le monde et qu'elle a mis à mal l'ensemble des structures de soins. C'est pourquoi les gouvernements ont été contraints de recourir au confinement pour limiter la propagation de la maladie et, ainsi, préserver les systèmes de soins d'un pic épidémique insoutenable pour nos organisations. Toutefois, les services vitaux pour la Nation ont maintenu leur activité : notre système de soins, évidemment, mais aussi, les premiers secours, les ambulanciers, les forces de sécurité, les personnels de l'éducation nationale, les crèches chargées d'accueillir les enfants des soignants, les services d'aide à domicile, les salariés des pompes funèbres, la grande distribution, la logistique. Les auteurs de cette proposition de loi estiment, à juste titre, que ces personnels ont été plus exposés que les autres à l'épidémie puisqu'ils ne pouvaient rester confinés, mis en arrêt maladie, en chômage partiel ou encore en télétravail. Ils estiment par ailleurs qu'une rupture d'égalité est apparue entre les soignants et les autres personnes mobilisées lorsque le ministre des solidarités et de la santé a annoncé que la Covid-19 serait reconnue comme maladie professionnelle pour les seuls soignants. Toutefois, concernant les autres travailleurs, monsieur le secrétaire d'État, vous avez annoncé le mardi 16 juin, lors d'une séance de questions d'actualité au Gouvernement, que lorsqu'ils ont été contaminés dans le cadre de leur activité professionnelle, ils pourront bénéficier d'une indemnisation au titre des maladies professionnelles. Vous avez également annoncé la publication, avec la ministre du travail, des décrets permettant cette évolution de la réglementation. Cependant, si cette mesure supprime la rupture d'égalité que nous évoquions précédemment, elle ne répond pas au champ de l'indemnisation prévue par le présent texte. En effet, comme l'a présenté notre En effet, comme l'a présenté notre collègue rapporteure Corinne Féret, que nous remercions de son excellent travail, les auteurs de cette proposition de loi ajoutent au forfait de prise en charge au titre des maladies professionnelles un principe de réparation intégrale des préjudices des personnes souffrant d'une maladie ou d'une pathologie consécutive à la contamination par la Covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l'exercice de leur profession ou d'une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l'être, ainsi que leurs ayants droit. Pour ce faire, ils proposent de créer un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19, géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en définissent son financement en créant une taxe additionnelle de 1,5 % à la taxe Gafam et en affectant une fraction des cotisations des employeurs à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Enfin, ils définissent la procédure de demande d'indemnisation auprès du fonds. Tel qu'il est présenté, ce texte nous invite à formuler plusieurs remarques. D'abord, il apparaît particulièrement difficile de caractériser l'origine de la contamination au SARS-CoV-2. En effet, cette maladie infectieuse se transmet par voie aérienne. Le docteur Élisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations au sein de la Haute Autorité de santé, professeure des universités à la faculté de médecine Xavier-Bichat et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, précisait notamment lors de la cinquantième journée Claude-Bernard en novembre 2007 que la transmission aérienne est définie par le passage de micro-organismes depuis une source à une personne à partir d'aérosols, entraînant une infection de la personne exposée. Elle ajoutait, d'une part, que, pour les petites particules, la transmission peut se faire jusqu'à une distance supérieure à 1,8 mètre et qu'un contact direct avec la source est inutile. Elle précisait que les maladies se transmettant par petites particules sont à l'origine d'épidémies brutales et explosives. d'autre part, que lorsque l'exposition s'opère par de grosses particules telles que des gouttelettes, il faut un contact proche, inférieur à 1 mètre. Pour les maladies ne se transmettant pas par petites particules, mais requérant des gouttelettes, la diffusion est lente, intermittente, variable et sans cluster. Enfin, si la contamination ne peut se faire que par contact direct avec les sécrétions respiratoires de la source, alors la transmission s'opère uniquement par le biais des sécrétions infectées depuis les mains jusqu'aux muqueuses respiratoires. En conclusion, en matière de maladies infectieuses, il est peu probable que nous puissions caractériser le lieu de la contamination. Ensuite, si nous n'ignorons pas que certaines personnes ont été mises en situation d'une surexposition, nous considérons qu'il ne faut pas confondre surexposition au danger du fait de son activité professionnelle et contraction de la maladie à l'occasion de la réalisation de cette activité. Présupposer qu'il y a eu contamination sur le lieu de travail paraît pour le moins particulièrement délicat en matière infectieuse, contrairement à l'exposition à l'amiante, dont le lien de causalité était certain et pouvait assurément être imputé à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Reconnaître ici cette fiction juridique revient par ailleurs à faire porter aux employeurs la charge symbolique de la responsabilité de la contamination de leurs employés. Or le lien de causalité entre activité professionnelle et contraction de la maladie ne pouvant pas être justifié, nous regrettons que la voie de la reconnaissance au titre des maladies professionnelles ait été privilégiée. J'ajoute que faire peser cette charge symbolique sur les employeurs privés, publics, ou sur les associations, alors que nous n'étions pas en capacité de leur permettre de protéger suffisamment leurs employés du fait de la pénurie de masques chirurgicaux et autres équipements de protection individuelle paraît d'autant plus injuste. C'est pourquoi, afin d'éviter toute différence de traitement entre les soignants et les autres professionnels mobilisés durant le confinement et afin d'éviter de faire porter aux employeurs la charge symbolique que je viens de décrire, je m'interroge sur le recours à une autre solution que le Gouvernement aurait peut-être pu privilégier plutôt que de faire porter cette charge par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Monsieur le secrétaire d'État, n'aurait-il pas été plus juste de garantir à ces travailleurs une prise en charge intégrale de la maladie, voire du préjudice, directement par l'assurance maladie sur présentation d'une attestation démontrant leur mobilisation durant le confinement ? C'est une réflexion. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera contre cette proposition de loi. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de nombreux travailleurs et bénévoles ont poursuivi leur activité professionnelle ou associative pendant le confinement mis en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19. professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, étaient sur le front, et l'ensemble des personnes mobilisées pour assurer la continuité de services essentiels à la vie de la Nation l'étaient également. Mais le manque de protections les a exposés à un risque accru d'infection. Certaines de ces personnes ont développé des formes graves de la Covid-19 qui ont pu donner lieu à une hospitalisation dans un service de réanimation, mais aussi à des atteintes respiratoires, neurologiques, cardiaques ou dermatologiques. Malheureusement, le pire s'est produit pour d'autres de ces professionnels, décédés des suites de cette contamination. Le texte soumis à notre examen ce matin par notre collègue Victoire Jasmin prévoit la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la Covid-19. Les auteurs de cette proposition de loi partent du principe qu'il appartient à la société dans son ensemble, et donc à l'État, d'assurer aux victimes de l'épidémie de Covid-19 une réparation simple, rapide et équitable de tous les préjudices subis. Nous avons tous été sollicités par des associations ou des fédérations professionnelles. En tant que rapporteure sur le suivi du Covid-19 en lien avec la branche assurance maladie, j'ai notamment auditionné des représentants de la Fédération de l'hospitalisation privée, qui m'ont également proposé l'organisation d'un dispositif juridique unique à l'échelon national destiné à indemniser les victimes du Covid-19. Je les remercie de leur contribution. Nous sommes très nombreux à avoir applaudi les soignants tous les soirs à vingt heures, sans pouvoir contribuer à la lutte contre cette épidémie sans précédent autrement qu'en restant chez nous. Aujourd'hui, nous ne pouvons que partager cet objectif visant à témoigner notre légitime reconnaissance, et celle de la Nation tout entière, aux personnels soignants qui se sont retrouvés en première ligne durant toute cette période, et à tous ceux qui ont pris en charge au quotidien nos concitoyens contaminés au cours des soins ou dans le cadre de l'organisation des soins de suite, et à tous les travailleurs et bénévoles, qui, au péril de leur vie, ont permis la continuité de secteurs prioritaires. L'article 1 de la proposition de loi définit les personnes potentiellement bénéficiaires. Le cadre est très large : il s'agit des personnes « souffrant d'une maladie ou d'une pathologie consécutive à la contamination par le Covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l'exercice de leur profession ou d'une activité bénévole, été en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées Les ayants droit sont également concernés. Les autres articles concernent, d'une part, la reconnaissance de la Covid comme maladie professionnelle et, d'autre part, la création d'un fonds d'indemnisation. Je salue votre travail, madame la rapporteure. Cependant, malgré les aménagements que vous aviez proposés lors de l'examen du texte en commission, le double dispositif continue à s'inscrire dans le cadre des maladies professionnelles. une reconnaissance en maladie professionnelle implique une prise en charge à 100 % des frais médicaux, des indemnités journalières majorées par rapport à un simple arrêt de travail et la possibilité d'une rente d'incapacité si les personnes gardent des séquelles. La mise en place d'un fonds d'indemnisation pour une contamination par une maladie infectieuse constituerait un précédent majeur qui bouleverserait les principes ayant jusqu'à présent prévalu pour engager la responsabilité de l'État et justifier d'une indemnisation.

Dériot, rapporteur de la branche AT-MP, « les maladies professionnelles sont établies en fonction des risques encourus dans le cadre d'une activité économique définie. Si l'on s'engage dans cette voie, nous créons un précédent pour les prochaines épidémies qui frapperont notre pays Cependant, nous saluons la mise en place du dispositif de reconnaissance automatique en maladie professionnelle de la contamination des soignants hospitaliers ou libéraux que vous avez présenté, monsieur le secrétaire d'État, dès lors que ceux-ci ont été exposés à un risque accru d'infection. Mais un risque accru en l'absence de matériel de protection suffisant, ce qui n'est pas sans poser la question de la responsabilité de cette absence de protection. Toutefois, cette proposition de loi va bien au-delà en instituant un principe de réparation intégrale des préjudices subis pour l'ensemble des personnes qui auraient exposé en milieu professionnel ou bénévole. Or, pour ces personnes, il sera particulièrement difficile d'établir l'origine professionnelle de leur contamination. L'adossement du fonds à l'Oniam, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, peu approprié. La vocation de l'Oniam, je le rappelle, est d'indemniser les dommages causés par un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale, une affection iatrogène liée à un traitement médical ou une infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé. D'ailleurs les associations et les fédérations proposant une indemnisation de ce type n'ont pas toutes la même approche. Si l'Association des accidentés de la vie, la Fnath, propose la création d'une commission d'indemnisation qui déterminerait les critères et les modalités d'accès à un fonds d'indemnisation déjà existant comme l'Oniam, d'autres, comme l'association Coronavictimes, demandé au Gouvernement de créer un fonds d'indemnisation des victimes du Covid-19 sur le modèle de celui des victimes de l'amiante, le FIVA, pour aller plus loin que la reconnaissance en maladie professionnelle.

a le mérite de s'attaquer à l'un des sujets de préoccupation des malades et de leurs familles. Toutefois, en proposant la création d'un fonds dédié à l'indemnisation rapide de toutes les victimes du coronavirus, les auteurs posent un certain nombre de questions aux législateurs que nous sommes, sans que la rédaction de la proposition de loi apporte, à notre sens, les réponses attendues. Car il s'agit bien ici de déroger au principe de la déclaration en maladie professionnelle pour une maladie infectieuse, ce qui constituerait une première et, pour certains, ouvrirait le risque à un champ de contentieux considérables. La reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles font l'objet d'un financement dédié à travers la branche AT-MP de l'assurance maladie et sont soumises à des critères stricts qui en garantissent une utilisation raisonnée et équitable. Ce mode de fonctionnement éprouvé permet aux victimes de maladie professionnelle de bénéficier de la gratuité des frais médicaux. En cas d'arrêt de travail, il leur donne accès à des indemnités versées par la sécurité sociale et l'employeur. En cas d'incapacité permanente de travail, une indemnité complémentaire leur est octroyée. Certes, ce système est loin d'être parfait. Une réflexion sur les réformes à envisager pourrait en effet être menée, afin de répondre aux critiques relatives à la complexité

tous les soignants et pour garantir aux non-soignants un accès à la procédure normale lorsqu'ils ont été contraints de travailler pour assurer la continuité de services essentiels à la vie de notre pays.

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous confirmer que, conformément à ce qui a été annoncé, tous les soignants bénéficieront de la reconnaissance en maladie professionnelle, y compris ceux qui n'ont pas cotisé pour le risque professionnel, ce qui est un sujet d'inquiétude sur le terrain ?

l'ai dit -, la création d'un fonds pour les victimes d'une maladie contagieuse ayant largement circulé dans la population créerait un précédent : nous devons faire preuve de prudence. Des maladies infectieuses apparaissent et disparaissent chaque année dans notre pays. Certes, la crise du Covid-19 a surpris par sa violence. Elle laissera des marques indélébiles en France et dans le monde entier. Néanmoins, une situation exceptionnelle n'appelle pas toujours des réponses exceptionnelles. Dans un premier temps, nous devons nous appuyer sur le système existant, quitte à l'adapter aux réalités cette crise sanitaire. Ce virus a fait de nombreuses victimes dans tous les pans de notre société. D'autres épidémies suivront probablement, hélas. Je suis donc convaincue que la création d'un tel fonds d'indemnisation ne répondrait pas totalement aux demandes légitimes de nos concitoyens ; en outre, elle ajouterait de la complexité. intéressés attendent, c'est surtout la mise en place d'un système performant, protecteur, équitable pour toutes les personnes exposées aux maladies professionnelles et qui ne laisse personne au bord du chemin. J'entends ceux qui invoquent la responsabilité de l'État pour justifier la création d'un fonds spécial.

ce cadre que des leçons pourront être tirées quant aux capacités de réaction de l'État. Si nous espérons qu'une crise de cette ampleur demeurera un phénomène exceptionnel, on ne peut pas oublier que l'augmentation des échanges internationaux, le réchauffement climatique et la mondialisation dans son ensemble provoqueront certainement de nouvelles épidémies. C'est en gardant cette réalité en tête que nous devons penser la prise en charge globale des victimes de maladies infectieuses dans le cadre de leur profession. Il y va de l'équité, valeur à laquelle nous sommes tous attachés.

de la maladie et sur la capacité d'adaptation du système à la crise que nous vivons. Ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement ont été davantage exposés à la contamination. Pour eux, un processus d'indemnisation plus simple et plus rapide doit être mis en place : c'est la volonté de l'État. Laissons

qu'ils soient professionnels ou bénévoles, et quel que soit le stade de l'épidémie de la Covid-19, a suscité l'émotion et l'admiration de tous. Dès l'apparition des premiers foyers de contamination sur le territoire de la République française, médecins urgentistes, infirmières en réanimation, personnels d'Ehpad ou même jeunes internes, tous se sont mobilisés pour prendre en charge les malades. À À cette occasion, ils ont été exposés à un risque parfois élevé de contamination. Bien au-delà du seul secteur du soin, de nombreuses personnes ont, tant bien que mal, maintenu leur activité pendant cette période afin d'assurer la permanence des services essentiels à la vie de la Nation. Je pense aux pompiers, aux ambulanciers, aux policiers et gendarmes, aux élus, aux enseignants chargés d'accueillir les enfants de soignants, aux aides à domicile, aux éboueurs, aux caissiers ou encore aux transporteurs routiers : qu'ils soient tous remerciés, et que ceux Parmi ces femmes et ces hommes, certains auraient développé des formes graves de la pathologie, pouvant entraîner des séquelles invalidantes ou incapacitantes- comme des atteintes respiratoires, cardiaques, dermatologiques ou neurologiques -ou provoquer des décès.

visant à « créer un fonds d'indemnisation spécifique pour les victimes de l'épidémie de Covid-19, qu'elles soient salariés du privé, fonctionnaires, indépendants ou bénévoles Ce texte comprend dix articles. L'article 1 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices des personnes souffrant d'une maladie ou d'une pathologie consécutive à la contamination par le virus et qui, préalablement à cette contamination, ont été, dans l'exercice de leur profession ou d'une activité bénévole sur le territoire de la République française, en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l'être, ainsi que ceux de crée un fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19, géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), le financement de ce

La contamination par le virus de la Covid-19 n'entre pas dans ce champ, et il serait inconcevable de créer un champ spécifique pour une maladie virale de ce type.

Cette règle s'appliquera aux soignants quels qu'ils soient et « quel que soit leur lieu d'exercice, à l'hôpital, en Ehpad ou en ville ». Les professionnels libéraux bénéficieraient eux aussi de ce mécanisme. Pour les autres travailleurs cités précédemment qui auraient pu être contaminés sur leur lieu de travail, il s'agira également de permettre une indemnisation au titre de la maladie professionnelle sans que celle-ci soit automatique. Cette reconnaissance sera mise en oeuvre dans les prochains jours, à la suite de la publication des décrets. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie d'en avoir clairement détaillé les modalités et de vous être engagé à agir au plus vite : c'est l'essentiel.

De même, lorsque la République rendra hommage aux victimes, il ne faudra pas oublier de citer les seize professionnels de santé décédés en essayant de sauver la vie des autres. étant, les personnels hospitaliers n'ont pas été les seuls à prendre des risques durant la pandémie en poursuivant leur activité. Il y a également les pompiers, les policiers, les caissières des magasins d'alimentation, les livreurs des plateformes, les égoutiers, les postiers, les éboueurs et l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui ont oeuvré pour le pays, eux aussi au péril de leur santé, parfois de leur vie. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour ces intérimaires envoyés en première ligne, souvent sans protection particulière, sans formation aux gestes de sécurité ou sanitaires,

Certaines de ces entreprises ont profité de la pandémie en réalisant un chiffre d'affaires exceptionnel tout en laissant leurs salariés sans dispositif de protection. L'enjeu est donc d'accorder reconnaissance et réparation à toutes les victimes de la Covid-19- salariés du privé, fonctionnaires, indépendants ou bénévoles, quel que soit leur statut -qui ont apporté leur aide dans la lutte contre l'épidémie et qui en gardent de graves séquelles. C'est l'objet de cette proposition de loi créant un fonds d'indemnisation spécifique pour l'ensemble des victimes de la Covid-19. Ce texte vise à trouver une solution face à une situation exceptionnelle,

Enfin, cette pandémie aveugle a touché à la fois des fonctionnaires, des salariés, des travailleurs indépendants et des bénévoles, catégories pour lesquelles les voies de reconnaissance des risques professionnels sont multiples. La solution préconisée par nos collègues socialistes afin de ne pas décourager les victimes d'une maladie qui n'entre pas dans les cases de notre système de réparation

comme la coordination des associations des victimes de l'amiante et de maladies professionnelles (Cavam), l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et autres maladies professionnelles (Andeva) et la Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés (Fnath).

dans le tableau de classification des maladies professionnelles, mais il a été jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, ce qui m'attriste. Selon nous, ce texte représente une avancée pour les victimes, même si nous avons quelques critiques à formuler.

outre, nous nous inquiétons du message potentiellement adressé au patronat, qui se plaint beaucoup de sa contribution à la branche accidents du travail-maladies professionnelles.

29 mars dernier, le Gouvernement a opté pour une reconnaissance au titre des maladies professionnelles pour tous les soignants malades du Covid-19. Cette reconnaissance donne accès à une couverture totale des frais médicaux, une indemnité d'incapacité de travail et, en cas de décès, à la perception d'une pension par les ayants droit. Cette règle s'appliquera aux soignants quel que soit leur lieu d'activité, à l'hôpital, en ville ou en Ehpad. Nous saluons cette annonce, mais nous comprenons les critiques qu'elle a suscitées. En effet, les soignants n'étaient pas les seuls à prendre des risques lors du confinement. Je pense notamment aux pompiers,

d'État, afin de compléter utilement ce dispositif, vous avez annoncé la semaine dernière que le Gouvernement allait étendre cette couverture à ces travailleurs qui se sont mobilisés pour assurer la continuité de leurs missions

qui n'étaient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale. Ces personnes ont pris des risques, pour elles-mêmes et pour leurs familles, dans des conditions d'hygiène et de sécurité parfois difficiles, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en masques de protection

dont on maîtrise mal les mécanismes, ne sera plus nécessaire, même si nos connaissances sur cette maladie restent imparfaites, notamment en ce qui concerne la grande diversité des symptômes et des séquelles associés.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi socialiste qui vise à réparer une profonde injustice. Nous souhaitons voir reconnaître et indemniser un préjudice, celui d'avoir été contaminé par le virus de la Covid en ayant permis à notre pays de vivre, lorsque la plupart d'entre nous se confinaient. Cette proposition de loi s'inscrit dans une continuité : le soutien aux victimes est défendu de longue date par les socialistes et par la gauche en général. Dernièrement, les travaux que le député de la Martinique Serge Letchimy a dédiés à l'indemnisation des victimes du chlordécone ont fait écho aux propositions d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques soutenues ici depuis 2012 par notre collègue Nicole Bonnefoy. Dans un autre domaine de risque, avec mon collègue Yannick Vaugrenard et bien d'autres, je soutiens régulièrement les démarches engagées par les associations de victimes de l'amiante pour une juste reconnaissance du préjudice subi. Je pourrais également citer les travaux en vue d'une juste indemnisation des catastrophes naturelles menés par Nelly Tocqueville ou pour une meilleure reconnaissance des victimes des essais nucléaires en métropole ou en Polynésie française.

ce député-ouvrier républicain socialiste obtint l'instauration, par la loi, d'une protection contre les accidents du travail. Il fut ainsi le précurseur de la branche AT-MP. le rapport de force qu'ils cherchent à rééquilibrer est souvent en défaveur des victimes. Si ces dernières sont nombreuses, leur indemnisation coûte cher et suscite des réserves et des précautions pour abonder les fonds.

La société dans son ensemble s'est montrée solidaire et une myriade de professions a contribué à « l'effort de guerre », pour reprendre les termes du Président de la République. À mon tour, j'en nomme quelques-unes : les hôtes et hôtesses de caisses de supermarchés et d'épiceries,

les éboueurs, toujours au rendez-vous, même quand le moindre emballage devenait suspect ; les conductrices et les conducteurs de transports en commun, confinés dans leurs cabines ; les membres des forces de l'ordre et de sécurité, les agents pénitentiaires, exposés sur le terrain, qui ont observé un régime de quatorzaines pour éviter de contaminer leurs unités ; l'ensemble des personnels des Ehpad, chargés des soins, de l'accompagnement, de l'entretien, des services de restauration et d'hébergement ou des tâches administratives

exhaustive. Mes chers collègues, il a fallu toute une nation pour faire face à cette pandémie et contenir sa propagation. Les personnes contaminées ont éprouvé la souffrance de la maladie, la détresse respiratoire, l'intubation, qui peut laisser des séquelles, et bien des symptômes. Après de longues semaines d'épuisement, certaines d'entre elles ont guéri, d'autres sont décédées. Ces personnes sont des victimes ; leurs proches et leurs ayants droit sont des victimes. Nous le reconnaissons pleinement et nous souhaitons les indemniser, parce qu'il serait injuste d'appauvrir davantage encore ces malades, qui ne sont en rien responsables de la pandémie. Bien qu'étant en deuxième ligne, ils étaient souvent les premiers et les premières de corvée. Tel est l'objet de cette proposition de loi, préparée par notre collègue Victoire Jasmin et construite avec l'appui du secteur associatif et des organisations syndicales. Saluons l'expertise

nous prévoyons que les connaissances scientifiques viennent compléter, par décret, l'appréciation de cette exposition et de ses conséquences devant

En commission des affaires sociales, les membres du groupe Les Républicains ont rejeté ces amendements, ce que nous regrettons. Je salue toutefois leur abstention constructive sur le texte, qui permet son examen en séance publique. Mes chers collègues, il n'est jamais trop tard pour bien faire

qui divise au lieu de rassembler semble loin d'être immédiatement efficace, y compris pour les professionnels de santé : faute de décret, les médecins libéraux qui ne cotisent pas à l'assurance facultative AVAT voient leur demande d'indemnisation rejetée.

pas à pas, comme cela a souvent été le cas pour les démarches d'indemnisation que j'ai citées au début de mon propos. Nous avons conscience que ce dispositif n'a pas vocation à répondre à tous les besoins, mais il vise large et n'instaure pas de tri : c'est là notre fierté.

et à limiter dans le temps le risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 rendant éligible au fonds une personne contaminée en milieu professionnel ou bénévole. bénévole. Les critères d'éligibilité prévus dans la rédaction initiale de l'article 1 ne sont pas opérationnels en pratique, compte tenu de l'impossibilité d'établir la réalité de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés. serait source de différences de traitement, et donc de contentieux. Il convient de poser les conditions d'une présomption irréfragable de contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole en définissant par une liste d'activités professionnelles ou bénévoles ayant exposé à un risque de contamination, étant précisé que cette liste ne saurait se limiter aux seules activités soignantes et qu'elle devra tenir compte du maintien en activité de secteurs publics ou privés d'importance vitale pour la Nation, que des critères objectivables permettant de présumer raisonnablement d'une contamination en milieu professionnel ou bénévole. Ces critères peuvent inclure la durée d'exposition au risque en milieu professionnel ou bénévole et, éventuellement, la liste des travaux exposant au risque. Ces éléments permettront d'organiser une procédure d'accès facilité à une indemnisation par le fonds, les victimes n'ayant plus à apporter la preuve de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés, ce qui est matériellement impossible. Il est prévu que le décret devant définir cette liste et ces critères devra

jeunes sont atteints par la Covid-19 parce qu'ils ont travaillé et livré des marchandises ou servi des gens, ils ne seront pas couverts. C'est à tous ceux-là qu'il faut penser ! Nous avons

prendra la forme d'une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances. Quel

est ainsi libellé : La parole est à M. Yves Daudigny. L'affectation d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale. Le troisième alinéa de l'article 7 de la proposition de loi, en ce qu'il prévoit l'affectation d'une partie du produit des cotisations AT-MP, est donc irrecevable au titre de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. vise à récrire cette disposition en prévoyant que le financement du fonds sera en partie assis sur une contribution de la branche AT-MP. Idéalement, il conviendrait que cette contribution soit prélevée sur les excédents cumulés depuis 2013 par la branche, afin d'éviter une augmentation de la part mutualisée des cotisations AT-MP. Quel

voix l'article 8. Mes chers collègues, je vous rappelle que si cet article n'est pas adopté, l'article 10 constituant le gage de la proposition de loi,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Mes chers collègues, les articles de la proposition de loi ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire. En conséquence, la proposition de loi, dans le texte